les réserves d’usage. Madame la ministre déléguée, mes chers collègues, depuis 2019, le 11 mars est la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme. C’est également la date choisie par l’Union européenne, en souvenir de l’attentat qui a eu lieu en 2004 à Madrid. Le terrorisme n’a pas de frontières. En cette journée de commémoration, nous pouvons nous souvenir des nombreuses victimes des actes de terrorisme qui ont ensanglanté à plusieurs reprises notre pays. Plus que jamais, nous devons rester unis face à cette menace et défendre les valeurs de la République. À la demande de M. le président du Sénat, je vous propose de commencer notre séance en observant une minute de recueillement en mémoire

la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc et de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, présentée par Mme Nadine Bellurot,

que Nadine Bellurot, Sonia de La Provôté, Didier Rambaud et moi même avons déposée en octobre 2024

Proposition de loi après proposition de loi, mission d’information après mission d’information, le constat de la crise de l’engagement local s’est imposé avec force, en particulier dans les communes rurales.

À l’issue du renouvellement général, 345 communes disposaient d’un conseil municipal incomplet. Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux qui avaient été observés en 2014, quand 74 communes étaient restées sans candidats et 228 sans conseil municipal complet.

Cette situation engendre pour les conseils municipaux des petites communes des difficultés de fonctionnement que chacun de nous ne connaît que trop bien. Les facteurs de crise des vocations électorales au niveau local sont multiples.

Nous sommes convaincus que les modalités du scrutin municipal qui s’appliquent dans les communes de moins de 1 000 habitants ne sont pas sans lien avec la démobilisation constatée et, plus généralement, avec les difficultés rencontrées.

Progressivement, le scrutin de liste proportionnel sans panachage ni vote préférentiel a été étendu à une part croissante des communes,

l’article 1 y autorise le dépôt de listes incomplètes. Seraient ainsi permis les dépôts de listes comportant au moins cinq candidats dans les communes de moins de 100 habitants,

La commission a souscrit à l’objectif principal de la proposition de loi et de la proposition de loi organique. Nous sommes convaincus en effet de la nécessité d’étendre le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants afin d’harmoniser les règles applicables

En plus de mieux protéger les maires, le scrutin de liste garantit la cohésion de l’équipe municipale autour d’un projet politique défini préalablement, là où le scrutin majoritaire contraint parfois le maire à constituer sur le tas, et de manière improvisée, une équipe visant à conduire la politique au au quotidien. Le scrutin proportionnel permet une expression du pluralisme politique, la diversité politique s’exprimant dans la liste.

troisième lieu, enfin, il semble difficilement concevable que les communes de moins de 1 000 habitants demeurent les seules collectivités à ne pas être concernées par le principe constitutionnel de parité.

et des présidents d’intercommunalité (AMF) et d’Intercommunalités de France, ont pris position en faveur de cette réforme. Comme nous, elles se disent convaincues du puissant levier qu’elle pourrait constituer pour enclencher une nouvelle dynamique au sein de l’engagement local. Il y a là un enjeu de vitalité démocratique pour les prochaines élections. Enfin, au sujet de l’entrée en vigueur des mesures proposées, il serait difficilement compréhensible que cette réforme ne s’applique pas dès l’année prochaine. Le retard dans le calendrier d’examen du texte n’est pas sans lien avec les soubresauts politiques des derniers mois. Je vous rappelle que la proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale voilà trois ans. En outre, l’article 28 de la loi Engagement et Proximité est ainsi

si le législateur a souhaité consacrer le principe de stabilité électorale, il a également admis la possibilité d’y déroger au cas par cas. En l’espèce, cette dérogation nous paraît totalement justifiée. Je rappelle, du reste, que l’élargissement

C’est pourquoi la commission a prévu des aménagements complémentaires de manière à garantir un dispositif opérationnel, suffisamment souple et adapté aux petites communes. Elle y est d’autant plus attentive que cette réforme a vocation à s’appliquer dès les prochaines élections municipales.

le sécuriser afin d’en assurer la pleine applicabilité et neutraliser les effets de bord qui pourraient résulter de la généralisation du scrutin de liste telle qu’elle est prévue par la proposition de loi initiale. Deux apports substantiels ont donc été introduits. En premier lieu, l’autorisation de déposer des listes incomplètes nous a semblé indispensable. Conçue dans un esprit de pragmatisme, cette dérogation est de nature à garantir le respect du pluralisme. Aussi la commission a t elle prévu

ou qu’il doit être complété en vue d’élire le maire ou plusieurs adjoints. Toutefois, ces élections auraient lieu au scrutin de liste, avec une plus grande souplesse pour le dépôt des listes. Si le principe est d’avoir des listes comportant le nombre de candidats nécessaire

cohérence avec l’ensemble de la réforme, la commission a par ailleurs procédé à deux harmonisations essentielles. La première consiste dans l’unification du mode de désignation des conseillers communautaires, grâce à

La seconde porte sur le mode de désignation des adjoints au maire. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints au maire seraient élus, comme c’est le cas dans les autres communes, au scrutin de liste paritaire. Toutefois, il est prévu une dérogation à la règle du remplacement de l’adjoint par un adjoint conseiller de même sexe, afin de répondre à la réalité de nos à la réalité de nos petites communes. En outre, la commission a souhaité répondre à une difficulté dont nous ont fait part les associations d’élus, et dont nous avions déjà à propos de l’application de la présomption de complétude en cas de vacance au sein du conseil intervenant postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection.

3, lever toute ambiguïté d’interprétation et permettre aux conseils qui se trouveraient dans cette situation de procéder directement à l’élection du nouveau maire, sans avoir au préalable

qui auraient pu résulter du texte adopté par l’Assemblée nationale. Elle a ainsi garanti, pour les communes de 500 à 999 habitants, le maintien du nombre actuel de délégués désignés au collège électoral des sénateurs, c’est à dire

qui démobilise nos élus locaux et nos maires, qui sont en première ligne. Dans nos petites communes, l’engagement des hommes comme des femmes est difficile ; il doit être facilité et encouragé. Cette réforme doit évidemment

la proposition de loi soumise à votre assemblée revêt une dimension démocratique non négligeable pour notre démocratie locale : il s’agit de garantir des règles électorales plus favorables à la constitution d’équipes cohérentes et moins fragiles, au service de toutes nos communes. Elle permet aussi d’œuvrer à une plus juste représentativité entre les hommes et les femmes. Ce texte privilégie le scrutin de liste et donne ainsi l’occasion de sortir du fameux panachage, lequel conduit trop souvent à des oppositions interpersonnelles parfois douloureuses au sein de conseils municipaux qui n’ont pas été constitués sur la base d’un projet partagé. Ce mode de désignation, appelé communément « tir aux pigeons », semble en effet de moins en moins accepté par ceux qui y sont soumis.

et se retrouvent ainsi placés dans une situation d’inconfort, voire de déstabilisation au quotidien. Le Gouvernement est bien évidemment conscient de ces difficultés, à l’heure où les vocations pour les mandats électoraux municipaux pourraient se tarir.

toutefois, chers sénateurs, qu’il peut être aussi difficile de trouver des colistiers que des colistières. N’oublions pas que, en milieu rural, les femmes sont souvent les premières engagées dans la vie sociale et associative des communes.

dont les conseils seraient réputés complets avec treize membres, pour un effectif légal de quinze conseillers. Ces dispositions majeures très attendues paraissent à même de garantir l’équilibre du texte, ainsi que le respect de l’exigence constitutionnelle de parité et d’expression pluraliste des opinions. À ce titre, puisque cette proposition de loi induit des adaptations du code électoral et qu’il est de la responsabilité du Gouvernement de sécuriser sur le plan juridique la tenue des élections municipales de 2026, le Conseil constitutionnel sera bien évidemment saisi. Si ce texte semble marquer une évolution significative,

force est de constater que cette réforme n’a pas compromis le fonctionnement de notre démocratie locale ni engendré de politisation particulière. Enfin, la parité dont il est ici question

la part des femmes parmi les élus locaux atteint près de 42 %, cette exigence d’une représentation équilibrée correspond également à une demande affirmée des associations d’élus locaux,

le sens profondément démocratique, ainsi que l’importance de cette proposition de loi. L’élection dans les 35 000 communes, dit elle, doit se faire « autour du triptyque “une commune, une liste, un projet” ». Au delà de cette question centrale du scrutin de liste, proposition de loi nous conduit également à examiner d’autres aspects de nos institutions locales. Sur les modalités d’élection des adjoints au maire, j’entends les arguments qui opposent les adversaires et les partisans d’une obligation paritaire. Je m’en remettrai, sur ce point, à la sagesse de votre assemblée.

un maire élu en cours de mandat à la suite de la démission de son prédécesseur pourrait en effet ne pas représenter sa commune à l’intercommunalité. Une telle situation constituerait un irritant et engendrerait des difficultés au sein d’une intercommunalité. Le Sénat et l’Assemblée nationale l’ont d’ailleurs admis en 2019,

Par ailleurs, des dispositions complémentaires sont prévues pour traiter la question de l’ajustement de l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles. À cette occasion, je souhaite saluer l’engagement de nombreux parlementaires au sein

L’ensemble des dispositions contenues dans cette proposition de loi ont vocation à entrer en vigueur à l’occasion de la prochaine échéance municipale de 2026. ou que c’est trop tard, mais sans doute est il tout simplement temps ! Enfin, cette proposition de loi est examinée conjointement à une proposition de loi organique qui tire les conséquences de la généralisation du scrutin de liste candidats ressortissants d’autres pays de l’Union européenne. Le Gouvernement est favorable aux évolutions proposées. Mesdames, messieurs les sénateurs, je le dis en conscience : ce texte est une nouvelle étape pour renforcer la démocratie locale et la rendre plus juste, mais aussi plus sûre. Il permettra de renforcer la cohérence des équipes municipales, de mieux protéger le maire, de consolider le fonctionnement de nos institutions

municipal soit bâtie autour d’un projet et d’une équipe. En conclusion, je veux remercier les rapporteurs et la commission de leur travail. Cette proposition de loi, qui suscite beaucoup d’attention, est le fruit d’un travail approfondi et d’une volonté transpartisane. Elle nous offre

ou des institutions immuables. Elle vit à travers celles et ceux qui s’engagent, à travers la diversité de nos élus, mais aussi à travers la capacité de nos collectivités à représenter la société. C’est dans ce même esprit de responsabilité et de dialogue

Pourquoi une telle précipitation à un an des élections municipales ? Pourquoi imposer un changement du mode de scrutin alors que les véritables urgences, comme la création d’un statut de l’élu local, sont laissées de côté ? A t on entendu les maires réclamer ce bouleversement ? Non Nos élus de terrain, ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps, très souvent bénévolement, pour le bien commun, demandent avant tout qu’on arrête de les noyer sous de nouvelles obligations et d’incessants changements des règles, qui ne répondent à aucun besoin exprimé par les territoires. Aucun ! Ils ne réclament rien d’autre

Plutôt que de les soutenir, on va leur ajouter, si nous adoptons ce texte, des contraintes inutiles et inadaptées. Les chiffres parlent d’eux mêmes : en 2020, plus de la moitié des maires ont eu du mal à constituer une équipe, 86 % d’entre eux ont peiné à trouver des volontaires, et 22 % ont affronté de graves difficultés pour respecter la parité.

Pourtant, c’est dans les communes de moins de 3 500 habitants que l’on trouve le pourcentage le plus élevé de femmes maires. Bravo ! Cette évolution s’est opérée sans contrainte, preuve que des dynamiques locales existent déjà. J’ai moi même été maire d’une commune de moins de 350 habitants. J’ai présenté une liste paritaire, sans y avoir été obligé, mais en convainquant simplement des personnes motivées, prêtes à servir leur commune, quel que soit leur sexe. Imposer des règles rigides de parité dans des villages où il est déjà difficile de trouver des volontaires, c’est méconnaître la réalité. Dans certaines petites communes, les habitants sont en majorité des hommes ; ailleurs, ce sont des femmes. Doit on refuser la candidature d’une personne motivée et disponible parce que l’équilibre entre les hommes et les femmes n’est pas atteint ? Quel non sens ! Plutôt que de modifier le mode de scrutin, ne devrions nous pas nous interroger sur les causes profondes de la crise de l’engagement municipal ? Au lieu de compliquer davantage la tâche des élus locaux, ne devrions nous pas concentrer nos efforts sur des réformes attendues, comme celles qui visent à renforcer la démocratie locale Il serait plus pertinent, par exemple, d’achever l’examen de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, qui répond aux véritables défis de reconnaissance et de valorisation du rôle de ces élus, et qui a été votée à l’unanimité au Sénat. derniers des moyens adaptés et un soutien institutionnel renforcé constituerait un levier bien plus pertinent pour encourager de nouvelles vocations et préserver la vitalité démocratique de nos territoires. Il faut qu’un élu puisse trouver un juste équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie privée et sa vie d’engagé au service de sa commune. C’était d’ailleurs la position de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales en octobre dernier, je me permets de le rappeler ! C’est faux ! Sa mission flash sur l’efficacité du fonctionnement des conseils municipaux

on a fait le bon diagnostic, on a dressé les bons constats, on a fixé des objectifs vertueux, mais on s’est perdu en route pour trouver des solutions, en imposant des règles stratosphériques sans tenir de compte des réalités de terrain et de la diversité des territoires Certes, cette réforme apporte des assouplissements, en réduisant le nombre de personnes requis pour constituer une liste ou en permettant de siéger dans un conseil municipal incomplet. Mais, pour le reste, elle ne fait que complexifier inutilement un système qui existe et fonctionne déjà bien.

est adopté, risque d’exacerber les tensions dans nos villages, où la solidarité et le vivre ensemble sont des piliers essentiels de la vie locale. Nous risquons de nous diriger vers une démocratie locale plus conflictuelle. Où est la fraternité ? On nous parle de « tir aux pigeons

Pis, nombreux seront les maires qui, face à cette complexité accrue, choisiront de renoncer. Le remède pourrait être pire que le mal ! Le danger ultime serait de voir des conseils municipaux disparaître faute de candidats, et nous savons tous où cela peut mener : à la disparation des communes

les textes que nous examinons aujourd’hui permettent de répondre à la préoccupation majeure que constitue la crise de l’engagement municipal, particulièrement dans les communes rurales de petite taille. Cette crise se manifeste partout en France

Afin d’enrayer cette spirale, il est nécessaire de faciliter l’engagement collectif dans tous les territoires et de créer les conditions de la cohésion municipale. Tels sont les enjeux de cette proposition de loi qui vise à étendre le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.

Les associations d’élus qui soutiennent cette initiative considèrent que le scrutin de liste peut favoriser l’esprit d’équipe, et donc l’engagement collectif et la réussite du projet municipal.

en évitant que les querelles de clocher ne se répercutent directement sur la vie démocratique. Ainsi, dans les communes de moins de 500 habitants, les conditions permettant au conseil municipal d’être réputé complet sont aussi assouplies. Enfin, l’obligation de parité reste souvent pour les maires des communes de petite taille un épouvantail, car elle est trop souvent contraignante, voire parfois injuste. C’est la raison pour laquelle il convient d’assouplir les effets de la parité sur l’équipe que constituent le maire et ses adjoints. le maire et ses adjoints. J’ai déposé un amendement visant à aménager le principe de parité lors de l’élection des adjoints dans les communes de moins de 1 000 habitants, afin de limiter ses contraintes pratiques pour les communes de petite taille.

Toujours dans cette logique d’adaptation au réel, il me semble nécessaire de protéger nos communes nouvelles. C’est tout le sens de mon amendement visant à prolonger la période transitoire au cours de laquelle les communes nouvelles bénéficient, à titre dérogatoire, d’un nombre de conseillers municipaux

C’est parce que la commune est la colonne vertébrale de notre confiance en la politique que notre démocratie locale doit être vivifiée pour être à la portée de tous. La parole Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un an avant les élections municipales de 2026, nous avons aujourd’hui l’occasion de légiférer sur deux sujets qui concernent de très près les élus locaux que nous représentons ici au Sénat : la parité et le mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants.

En effet, lors de nos travaux, nous avons constaté que les femmes ne représentent que 37,6 % des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, contre 48,5 % dans les communes de 1 000 habitants et plus. Ces communes de moins de 1 000 habitants constituent pourtant 71 % des communes françaises. Dans la mesure où les modes de scrutin sont actuellement différents selon la taille des communes, une harmonisation aurait donc inévitablement pour effet d’augmenter le pourcentage de femmes exerçant des fonctions électives au sein du bloc communal. J’ajoute par ailleurs que ce renforcement de la parité dans les communes pourrait aussi, par voie de conséquence, entraîner une meilleure représentation des femmes dans notre assemblée sénatoriale. Ensuite, je considère que l’harmonisation des modes de scrutin pourrait avoir d’autres avantages. Le scrutin de liste favorise la constitution des équipes et l’émergence d’un collectif, qui ne se résume pas à l’addition d’intérêts particuliers.

Dans les villages, là où la personnification de l’élection est particulièrement puissante, cela peut, à mon avis, desservir notre démocratie locale. En transformant le scrutin majoritaire en scrutin de liste paritaire, nous inciterons demain les citoyens à voter pour des projets et non pas contre des candidats. On connaît, hélas ! le sort réservé à certains élus sortants qui n’auraient pas accordé, ici ou là, quelques autorisations d’urbanisme,

Enfin, je voterai pour l’adoption de ces textes, car ils permettront d’instaurer de nouveaux mécanismes de souplesse, adaptés aux réalités électorales.

de moins de 1 000 habitants, ou encore aux règles de désignation des adjoints au maire. Mes chers collègues, je comprends que ces sujets puissent être source de débat. J’ai échangé, comme chacun de vous, avec de nombreux maires de mon département, et je sais que leurs avis sont partagés. Néanmoins, je voudrais insister sur le communiqué de presse des associations nationales d’élus locaux publié le 6 février dernier. Ce communiqué est très clair : il indique que ces associations soutiennent, depuis 2020, l’instauration du scrutin de liste dans toutes les communes, y compris pour les élections municipales de 2026.

le 8 juillet dernier, nous célébrions le vingt cinquième anniversaire de la révision constitutionnelle relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. Celle ci posait ce principe simple, mais indispensable : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Cette réforme a ainsi permis de prendre par la suite des mesures législatives pour améliorer la parité parmi les représentants politiques.

Ce combat pour instaurer la parité parmi les élus locaux doit faire consensus, car c’est le corollaire de la promesse républicaine et démocratique. Ce préalable étant posé, j’en viens à la question des modalités de scrutin permettant d’atteindre l’objectif de parité. Cette problématique se double d’un constat contemporain et largement admis d’une crise de l’engagement local dans les communes rurales. Le nombre de candidats à des fonctions municipales baisse et, en octobre 2024, Ces chiffres doivent nous alarmer et nous conduire à légiférer. Ainsi, pour répondre à l’objectif constitutionnel de parité ainsi qu’à cette crise, le choix est fait, dans ce texte, d’appliquer le scrutin proportionnel et paritaire de liste à toutes les communes. Cette solution s’inscrit dans la continuité des réformes précédentes du droit électoral. Le passage à ce mode de scrutin emportera nécessairement des conséquences majeures sur les modalités des campagnes politiques dans les communes concernées.

de protéger la cohésion des équipes municipales des effets pervers du scrutin majoritaire préférentiel avec panachage. Je regrette toutefois que les délais imposés par les prochaines

nous examinons, la commission des lois a souhaité valider le principe de l’harmonisation du mode de scrutin entre toutes les communes, tout en sécurisant le dispositif. Je tiens à saluer le travail de nos rapporteurs, qui ont intégré une certaine souplesse dans l’application de la loi, notamment pour favoriser le pluralisme.

Dans tous les cas, nous assurons collectivement de notre soutien les élus des communes rurales, qui témoignent au quotidien de leur engagement démocratique en faveur de l’intérêt général.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comment encourager l’engagement dans nos communes, dans ces « petite[s] république[s] dans la grande », comme le rappelle souvent le président du Sénat, faisant siens les mots de Jules Barni ? C’est en somme la question à laquelle ces deux textes visent à répondre. Commençons par un constat sans appel : en 2020, après les élections municipales,

une partie de la solution, laquelle ne pourra être complète que si l’on apporte plusieurs améliorations au fonctionnement des conseils municipaux, dans la perspective des élections municipales de 2026.

provient de nos collègues de l’Assemblée nationale, qui ont également apporté leur pierre à cet édifice collectif. Quelles sont donc les améliorations

Permettez moi de saluer l’excellent travail de nos rapporteurs, Nadine Bellurot et Éric Kerrouche, qui ont proposé à la commission des lois d’adopter des amendements, afin de sécuriser le texte pour nos plus petites communes. Car c’est bien là

Il restera un sujet à traiter, madame la ministre, qui est évoqué sur toutes les travées : il s’agit du nombre d’élus dans les conseils municipaux et de sa possible réduction. Cette proposition de loi lance le débat

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à rappeler que notre groupe a toujours défendu la parité. Je souhaite d’ailleurs rendre hommage à la présidente Hélène Luc, qui, en 1999,

la proposition de loi et la proposition de loi organique que nous devons examiner aujourd’hui ne se cantonnent pas à la question de la parité et portent plus largement sur l’instauration du scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants. L’objectif, plus que légitime, de la parité, mis en avant par les auteurs des textes, est donc subordonné à la modification du mode de scrutin. Or, mes chers collègues, si le scrutin de liste semble désormais adapté aux communes de plus de 1 000 habitants,

Alors que la crise de l’engagement local nous préoccupe tous, que 5 % des maires ont démissionné depuis 2020, et que les prochaines élections municipales sont dans un an, toute modification du mode de scrutin doit être faite avec minutie.

La technique de panachage qui existe aujourd’hui donne aux électeurs la possibilité de construire eux mêmes la liste qui les représentera le mieux. Quel modèle de démocratie ! Les élus n’ont alors d’autre choix que d’avancer ensemble, selon la volonté de leurs électeurs. L’absence de prime majoritaire favorise en plus

pour que leur engagement soit réellement soutenu. Or la modification du mode de scrutin semble aller à l’encontre de cet objectif. La crise de l’engagement est le défi majeur qui

l’inscription à l’ordre du jour de ces deux textes, qui visent à mettre fin au mode de scrutin plurinominal majoritaire avec possibilité de panachage, est vraiment – vraiment ! – une bonne nouvelle pour la démocratie locale. Proposer aux citoyens de barrer certains noms est devenu totalement anachronique aujourd’hui. Le panachage faisait ressortir les comportements les plus éloignés des valeurs républicaines : misogynie, racisme, intérêts particuliers. J’ai vu, comme maire, des bulletins où les noms de colistiers ou colistières à consonance étrangère étaient barrés. C’est une réalité. Souvent, et nous l’avons tous constaté, le maire ou l’adjoint à l’urbanisme est sanctionné pour avoir défendu l’intérêt général. La discussion de ces textes est finalement l’aboutissement de la réforme de 2013, qui avait instauré le scrutin de liste proportionnel pour les communes entre 1 000 et 3 500 habitants. Depuis la révision constitutionnelle de 1999, nous avons progressé dans la garantie de l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. La parité est atteinte dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux et dans les communes de plus de 1 000 habitants. Le combat n’est pourtant pas gagné. Sur le plan quantitatif d’abord : le Sénat et l’Assemblée nationale comptent à peine plus d’un tiers de parlementaires femmes, alors que, pour la Chambre haute, le scrutin de liste devrait réduire significativement la part d’hommes sur nos travées ; nous comptons 37,5 % de conseillères municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, et je ne parle pas des intercommunalités. Sur le plan qualitatif, ensuite : la sociologie, qui renseigne assez précisément la répartition genrée des postes au sein des exécutifs, montre que les femmes sont le plus souvent cantonnées aux secteurs intéressant moins les hommes, car perçus comme des champs secondaires L’évolution du mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants est un palier supplémentaire vers une meilleure représentation des femmes dans l’ensemble des conseils municipaux. À chaque palier, nous avons trouvé des détracteurs pour dire, au mieux,

aux collectivités territoriales du Sénat, et a été déposé en octobre 2024. Comme cosignataire de la proposition de loi organique de M. Kerrouche, je soutiens évidemment cette évolution du droit. Le calendrier n’est cependant pas sans poser des difficultés. Alors que nous discutons de dizaines de propositions de loi au Sénat par session, il faut attendre à peine douze mois avant l’échéance que nous nous prononcions sur ce sujet. La proposition de loi organique, non encore examinée par l’Assemblée nationale, va devoir l’être en première lecture, avant une éventuelle CMP. Je dis « éventuelle », puisque le Gouvernement n’a pour l’heure toujours pas déclenché la procédure accélérée. Pour autant, madame la ministre, je tiens à saluer votre ténacité ténacité sur ce sujet. Encore une fois, nous subissons un manque d’anticipation et nous légiférons à la hâte, avec un impact évident pour la constitution des listes de candidates et candidats déjà en cours pour les communes de moins de 1 000 habitants, qui représentent tout de même tout de même 73 % des communes. Nous saluons le travail fait par la commission des lois pour faire cheminer le texte à partir de la version issue des travaux de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat. Ce texte est plus équilibré, parce qu’il ne se résigne pas réduire le nombre d’élus. Plus que jamais, face aux défis de notre époque, les petites communes ont besoin de citoyens engagés au sein de leur conseil pour assurer la charge publique locale toujours croissante. Il convient également d’avancer sur le statut de l’élu, sans oublier le cas des élus municipaux sans délégation, pour lever les freins à l’engagement et lutter contre le découragement.

ces propositions de loi s’attaquent à l’une des résistances structurelles et persistantes de notre démocratie locale, à savoir la différenciation des modes de scrutin. Je tiens, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à saluer le travail accompli par nos deux collègues rapporteurs, Nadine Bellurot et Éric Kerrouche. Ce sujet nous a naturellement mobilisés de manière transpartisane.

l’AMRF, l’AMF et Intercommunalités de France. Aujourd’hui, le Sénat, représentant de nos communes, a une responsabilité historique

Car, oui, l’égal accès aux mandats locaux est non pas une option, mais une exigence républicaine. Le cœur de ce texte est la généralisation du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Cette mesure, qui s’appliquerait à près de 70 % des communes françaises, constitue une réponse pragmatique et efficace pour favoriser l’émergence d’un vivier de candidatures. Loin d’être une contrainte, cette évolution permettra notamment de faire en sorte que l’engagement des femmes ne soit plus une exception. En instaurant un scrutin de liste paritaire, nous encourageons les citoyens à présenter des candidatures mixtes. C’est une avancée concrète qui s’inscrit dans la continuité des lois adoptées ces vingt dernières années. La commission a apporté des améliorations significatives au texte initial, tout en conservant son ambition première. Ces ajustements visent à garantir l’opérationnalité juridique du dispositif et témoignent d’une volonté de répondre aux réalités du terrain. Ce texte introduit ainsi une marge de manœuvre pour les communes comptant entre 500 et 999 habitants, dont les listes pourront être considérées comme complètes si elles comptent treize candidats au lieu de quinze. Cet ajustement progressif facilite la mise en œuvre du scrutin de liste sans alourdir les contraintes pesant sur ces communes ni créer de nouveaux seuils administratifs inutiles. Cela permet aux petites communes de fonctionner normalement même si leur conseil municipal n’est pas complet, réduisant ainsi les contraintes administratives et les coûts liés aux élections complémentaires. autant, la commission a souhaité que les communes de 500 à 999 habitants conservent le même nombre de délégués au collège électoral des sénateurs, c’est à dire trois, quand bien même elles compteraient treize conseillers municipaux au lieu de quinze. Nous remercions la commission d’avoir veillé à neutraliser les éventuels effets indésirables Nous saluons également le maintien du mécanisme d’élections complémentaires pour les communes de moins de 1 000 habitants, lesquelles auraient lieu au scrutin de liste paritaire. Ces scrutins bénéficieraient des mêmes souplesses que celles qui sont prévues pour les renouvellements généraux, à savoir la possibilité pour les listes de compter deux candidats en moins ou deux candidats en plus que le nombre de sièges à pourvoir. L’objectif est clair éviter la multiplication des élections partielles intégrales et préserver la stabilité des conseils municipaux. Toujours dans cette logique d’adaptation à la diversité de nos communes, mon groupe a déposé un amendement visant à proroger le système dérogatoire relatif à l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles jusqu’au second renouvellement général. Ce dispositif répond à une réalité simple les communes nouvelles, souvent issues de fusions récentes, ont besoin de temps pour trouver leur équilibre et construire une dynamique collective. En étendant la période de transition, nous leur offririons la possibilité de s’organiser pleinement, tout en garantissant une meilleure représentation des communes déléguées au sein des conseils municipaux. Cette mesure est pragmatique et témoigne de notre volonté de soutenir les territoires dans leur diversité, de respecter leurs rythmes et de leur donner les moyens de réussir leur transformation. En ce qui concerne l’harmonisation du mode de désignation des adjoints au maire, l’application du scrutin de liste paritaire aux plus petites communes répond à l’ambition générale de ce texte. Cette évolution ne remet pas en cause l’organisation, puisque, en cas de démission ou d’empêchement d’un adjoint, son remplacement pourra s’effectuer sans contrainte de sexe.

la représentation des femmes dans les exécutifs intercommunaux, mais nous entendons surtout la volonté d’accorder la priorité aux communes de moins de 1 000 habitants dans ce texte. À l’approche des élections municipales de 2026, la crise de l’engagement local demeure une réalité préoccupante, particulièrement dans nos petites communes. La crise des vocations, que nous observons tous depuis plusieurs années et qui fait l’objet de nombreux débats dans n’est pas une fatalité : elle est le symptôme d’un désenchantement et d’un épuisement face à des mandats devenus trop lourds, trop exposés et qui sont trop peu reconnus. Comme le souligne le rapport, cette crise se manifeste par une baisse alarmante du nombre de candidats et une augmentation sans précédent des démissions en cours de mandat. En 2020, 345 communes ne disposaient pas d’un conseil municipal complet, et plus de 5 % des maires élus cette année là avaient démissionné au 1 octobre 2024. Ces chiffres illustrent une situation critique qui menace à la fois la stabilité et le fonctionnement de nos institutions locales, fragilisant nos territoires. Face à cette réalité, il est urgent de redonner du sens et de l’attractivité à l’engagement local. Ce texte, en généralisant le scrutin de liste paritaire pour les communes de moins de 1 000

En instaurant un scrutin de liste, nous encourageons la constitution d’équipes municipales plus soudées autour d’un projet politique commun et nous brisons le plafond de verre qui empêche les femmes de s’engager pleinement dans la vie politique locale, tout en mettant fin fin à la pratique du « tir aux pigeons », qui fragilise souvent les maires et déstabilise les conseils municipaux dans le temps. Pour toutes ces raisons, c’est avec la conviction

Au printemps puis à l’automne 1945, lors des élections municipales et législatives, nos aïeules découvraient ces droits civiques jusqu’alors réservés à la mâle assemblée : le vote et l’éligibilité. Elles furent ainsi un peu plus de deux cents à devenir maires, et trente trois à entrer à l’Assemblée nationale Depuis lors, société et législation ont évolué. Les femmes exercent désormais plus de responsabilités, notamment politiques, et le pays ne s’en porte pas plus mal. Sans vouloir faire de la psychanalyse de comptoir, je dirai que la complémentarité entre Mars et Vénus n’est pas une caricature. La loi a eu un rôle clé pour esquisser une meilleure représentativité du personnel politique et l’objectif de parité doit être salué. Néanmoins, bien légiférer, c’est à dire rendre possible ce qui est souhaitable, n’est pas toujours aisé. Si certains textes s’avèrent quasi parfaits – je pense à l’instauration des binômes dans les cantons de nos départements –, certaines bonnes intentions peuvent se révéler fâcheuses. La loi, jusqu’à présent, a considéré que les communes de moins de 1 000 habitants devaient bénéficier d’un processus électoral particulier. Le texte dont nous débattons reviendrait à appliquer désormais aux 34 871 communes de France exactement les mêmes modalités de scrutin. Il s’agirait donc d’imposer aux 25 000 villages de moins de 1 000 habitants l’obligation de présentation de listes paritaires. Or, si la règle n’est pas la même pour tous, c’est non pas par hasard, mais parce que le législateur a considéré qu’il était trop difficile d’appliquer le principe de liste paritaire dans nos petites communes. Non pas que les ruraux soient rétifs à avoir des femmes pour édile. Bien au contraire ! Le pourcentage de femmes maires d’une commune de moins de 1 000 habitants est ainsi supérieur à celui des cités plus peuplées. C’est la constitution de la liste qui pose problème. Et par ces temps mauvais de désengagement républicain, de fonte des glaces citoyennes, personne ne peut nier que la quête de candidats et de candidates relève du chemin de croix. Est il pertinent aujourd’hui d’instaurer une contrainte supplémentaire, fût elle vertueuse, pour bâtir nos conseils municipaux ? J’ai interrogé par sondage les élus des 680 communes de l’Oise, parmi lesquelles 500 comptent moins de 1 000 habitants. Le résultat est net les deux tiers des élus sont défavorables à cette mesure. Voici quelques unes de leurs réflexions. Christine Ortegat, maire de La Neuville sur Oudeuil : « J’y suis favorable, mais je peine à trouver ou à motiver des candidates. La parité obligatoire me semble un obstacle pour constituer une équipe solide. » Pascal Wawrin, maire de Villers Saint Sépulcre Aujourd’hui, trouver des administrées qui souhaitent s’impliquer est compliqué ! La parité ajoute une pression supplémentaire, dans un contexte difficile, et peut finir par décourager. Carole Gautier, maire de Senots : « Il n’est pas envisageable de remplir une liste avec des noms simplement pour répondre à une règle de parité. La seule règle est le volontariat et celui ci n’est pas genré.

parmi les sortants désirant poursuivre leur mission municipale, des élus compétents et investis uniquement parce qu’ils sont du mauvais genre. Dommage pour celui ou celle qui, depuis des années, consacre son énergie à la commune et qui devra peut être céder sa place à quelqu’un de moins motivé, mais avec le bon chromosome. Cela est il juste ? si la parité obligatoire a une vocation de juste représentativité, nos conseils paritaires deviendront ils le miroir idéal de la société ? N’y aurait il pas trop de retraités ? Pas assez de jeunes ? Où doit s’arrêter la logique des quotas ? N’ouvre t on pas la boîte de Pandore ? Confondant volontarisme et aveuglement, niant la réalité avec une vision idéalisée et idéologique, cette loi risque de mettre à mal de nombreux conseils municipaux et de fragiliser toute la ruralité. Je ne voterai donc pas ce texte à la teinte de miel, mais à la saveur de fiel.

les textes que nous étudions cet après midi représentent, de mon point de vue, une triple avancée : démocratique, politique et sociale. Avancée démocratique, tout d’abord,

tous nos concitoyens pourront élire leurs conseillers municipaux dans les mêmes conditions électorales, quelle que soit la strate de population de la commune concernée. Avancée politique, ensuite, car le scrutin proportionnel pour une élection locale permet de constituer une réelle dynamique d’équipe au service de projets de proximité.

Ce choix permet aussi la représentation des minorités et favorise donc la participation d’un plus grand nombre de citoyens au choix de ses représentants municipaux. Il reprend d’ailleurs la recommandation n° 64 du rapport, dont j’avais dont j’avais été le corapporteur en 2021 avec d’autres collègues de la délégation aux droits des femmes. Avancée sociale, enfin, car l’extension du scrutin de liste s’accompagne de l’obligation de parité.

La parité est un moteur de l’engagement des femmes dans la vie politique locale et n’est en aucun cas, comme j’ai pu l’entendre encore ce soir, une contrainte administrative ou, pis, une menace pour l’existence des communes rurales. J’entends souvent également que le faible nombre d’habitants dans les communes concernées, en majorité dans les espaces ruraux, pourrait rendre complexe la mise en place de ce scrutin. Pourtant, en 2021, le rapport de la délégation aux droits des femmes auquel je faisais allusion

La société, me semble t il, est mûre. Elle le prouve déjà aujourd’hui en votant pour des maires qui sont des femmes et en votant pour des sénatrices, pour des députées. Il faut maintenant que nous puissions aller au bout pour toutes les communes.

aller plus loin que l’esquisse d’une parité et faciliter leur engagement sans faire la révolution ni martyriser les hommes. Et chacun sait que, dans ma vie de sénatrice, je n’étais pas connue pour être

J’ai effectué une visite officielle dans vingt six départements. Quand je me déplace, je ne vais ni dans les métropoles ni dans les grandes villes. Les gens me parlent avec spontanéité : quand ils ont envie de me dire des choses désagréables, ils le font.

à partager la volonté d’harmoniser le mode de scrutin, de supprimer le système ancestral du panachage, de mettre en place un scrutin de liste et d’autoriser le dépôt de listes incomplètes, il en va tout autrement en ce qui concerne la contrainte paritaire que prévoit l’article nous savons mieux que quiconque la difficulté que peut représenter la constitution d’une équipe municipale dans nos petites communes. Trouver des volontaires pour s’engager est déjà un défi. Compétence, disponibilité, motivation, sens de l’engagement : voilà des critères légitimes pour choisir ces colistiers. Ajouter un critère de répartition artificielle, c’est prendre le risque d’écarter des candidatures précieuses, faute de respect du quota imposé. Pis encore, c’est augmenter le risque de listes incomplètes. Faisons confiance à nos élus et à nos concitoyens. Cet article repose sur une idée partiellement fausse. En effet, la proportion de femmes maires est plus forte dans les petites communes qui n’ont pas d’obligations paritaires que dans les grandes. l’échelon national, plus de 21 % des maires de commune rurale sont des femmes, contre moins de 18 % dans les communes urbaines. L’engagement féminin doit se construire par la légitimité démocratique, non par la contrainte

Je ne peux que vous encourager aujourd’hui à la même réserve et à ne pas toucher à l’équilibre actuel. Oui ! Ce texte risque en effet de créer bien plus de difficultés qu’il n’est censé en résoudre. Dois je vous rappeler que nous ne cessons de déplorer la crise de l’engagement municipal ? Croyez vous qu’imposer des contraintes supplémentaires aux petites communes les aidera à attirer des candidats ?

Pourquoi ne pas prendre en compte d’abord la motivation ? Cette parité au forceps n’est ni avisée ni respectueuse des attentes locales.

à plus long terme, comment ne pas y voir une pression déguisée vers les regroupements forcés de communes ? Eh oui ! Pour finir, la commission souhaite promouvoir la cohésion de l’équipe municipale autour d’un projet politique avec le scrutin Je crains que ce vœu de remobilisation politique, certes louable, ne se révèle finalement clivant et très inadapté au quotidien des très petites communes, où les bonnes volontés se fédèrent autour de projets concrets.,

nous pouvons reconnaître qu’en France nous ne sommes pas les plus audacieux pour faire progresser les droits des femmes et la parité. Les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1945 le droit à un compte bancaire qu’en 1965. Bien plus, le port du pantalon a été officiellement reconnu en 2013. Sur la question de la parité dans les élections municipales, je salue le large consensus de toutes les associations d’élus, qui y sont progressivement devenues favorables. Pour

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre pays traverse une véritable crise de l’engagement local. Dans nos villages et nos petites communes, les vocations d’élu municipal se font de plus en plus rares. Accablés par des responsabilités croissantes, des contraintes administratives toujours plus lourdes et un manque criant de soutien, ces élus, pourtant indispensables à la vie de nos territoires, renoncent. Ce problème n’est pas anodin. Il est le symptôme d’un pouvoir central qui, au lieu de renforcer la démocratie locale, l’étouffe sous des réformes déconnectées des réalités du terrain. L’article 1 s’inscrit dans cette logique en imposant un scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants. Il vient complexifier encore davantage la vie municipale. Jadis, dans ces petites communes, on votait avant tout pour des personnes, pour des citoyens engagés au service de leurs voisins. Ce système garantissait une démocratie vivante. Désormais, en imposant un scrutin de liste avec une logique paritaire, on contraint ces communes à adopter une logique partisane qui va complexifier les élections et freiner l’engagement de nombreux citoyens. Que dire de la complexité introduite par ce texte ? On nous parle de listes complètes, de seuils de candidats, d’élections complémentaires soumises à de nouvelles règles : c’est un véritable casse tête pour des communes qui, vous le savez, mes chers collègues, peinent déjà à mobiliser des volontaires. La ruralité n’a pas besoin d’une nouvelle contrainte administrative ; elle a besoin de liberté et de simplicité. Dans de nombreuses petites communes, il est déjà difficile de trouver des élus motivés. Désormais, avec ces nouvelles obligations, nous risquons de nous retrouver avec des élections impossibles à organiser et des conseils municipaux dysfonctionnels. Le Rassemblement national, fidèle à sa défense des territoires et de la proximité entre les élus et les citoyens, refuse cette réforme qui éloigne encore un peu plus les Français du pouvoir local. Ce texte ne répond à aucune demande des élus de terrain et ne fait que complexifier une organisation qui fonctionnait jusqu’à présent. Plutôt que d’imposer un modèle pensé pour les grandes villes, nous devons au contraire protéger nos petites communes, leur offrir plus de souplesse et encourager l’engagement citoyen. Nous voterons donc contre l’article 1, car nous croyons en la démocratie locale, en la souveraineté des communes et en la voix des Français, qui refusent qu’on leur impose un modèle uniformisé. La France des territoires ne doit pas être sacrifiée sur l’autel d’une centralisation toujours plus pesante. Nous défendrons toujours nos villages, nos élus locaux et l’esprit démocratique qui les anime. La parole

à ces maires qui veulent le scrutin de liste, mais pas la parité ? À ceux qui veulent la parité, mais pas le scrutin de liste ? À ceux qui veulent bien réduire les effectifs des conseils municipaux, à condition que

Je voudrais que le Sénat perde l’habitude de cultiver l’art de répondre à des questions qui ne lui sont pas posées. Aujourd’hui, les élus ne nous demandent

moyens et la fin des incivilités, voire des agressions dont ils sont victimes. En bref, ils ont besoin d’être soutenus. À la veille des élections municipales,

? Dans les communes de moins de 1 000 habitants, on constitue des équipes et on fait en sorte qu’elles soient représentatives. Bien entendu, nous défendons tous la parité, mais, ce que nous défendons surtout, c’est la représentativité dans notre territoire des différents hameaux, des différentes professions, des différentes sensibilités qui feront que l’acte démocratique sera que l’acte démocratique sera au rendez vous. À mon sens, non seulement le Sénat perd son temps, mais il est de surcroît en train de perdre son âme. Nous sommes les représentants des territoires, les représentants de ces petites collectivités. À force de réduire le nombre d’élus

ce vers quoi on tend quand on a la responsabilité d’une commune. Un projet commun promu par une équipe qui a été élue est un gage de transparence, une forme de loyauté vis à vis des électeurs qui ne connaîtront ni surprise ni imprévu. C’est une forme d’efficacité

pourquoi y aurait il des difficultés à avoir autant de femmes que d’hommes dans un conseil municipal ? Pourquoi y aurait il plus de difficultés dans une commune de petite taille ou de très petite taille ?

Mais enfin, pourquoi le Gouvernement s’attache t il aujourd’hui à faire la guerre à la liberté ? Oui, la liberté de choisir librement ceux que l’on veut élire.

Le scrutin est ouvert.

le monde des collectivités locales, singulièrement celui des communes, n’est pas un ensemble homogène. Il existe des différences importantes entre les très grandes villes, les grandes villes et les tout petits villages, qui comptent parfois moins de dix habitants.

norme. Je propose donc de réserver la possibilité de déposer des listes incomplètes aux communes de moins de 500 habitants, qui, dans les faits, disposent d’un gisement plus faible de candidats.

la désignation des conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau comme conseillers communautaires. C’est un sujet sur lequel

chacun son choix

Quel est l’avis de la commission ?

l’avis du Gouvernement

Il s’agit d’un amendement de simplification au bénéfice des communes nouvelles, puisqu’il vise à prolonger la période transitoire au cours de laquelle ces communes bénéficient de règles dérogatoires

historiques ». Cette interprétation pose des difficultés très concrètes, puisqu’elle contraint, si le conseil municipal a perdu plus du tiers de ses membres, à organiser le renouvellement intégral du conseil pour procéder à l’élection d’un nouveau maire ou de nouveaux Or qui dit renouvellement intégral dit fin de la période transitoire et, partant, basculement dans le droit commun pour la commune nouvelle. Nous avions déjà identifié de telles difficultés, puisqu’une proposition de loi d’origine

Madame Bourcier,

de conserver la proximité et la représentativité nécessaires, un mandat supplémentaire avec un effectif supérieur ne sera pas de trop. Enfin, il est nécessaire de prendre en compte le fait que nombre de communes nouvelles n’ont que dix ans d’existence et qu’elles ont besoin d’équipes solides pour monter en compétence et faire face à de telles mutations. Le sous amendement

Le code général des collectivités territoriales prévoit ainsi, lors du second renouvellement général, un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. La crainte est donc forte que, avec cette baisse brutale des effectifs, les communes historiques ne soient pas suffisamment représentées. Cela est d’autant plus vrai pour les communes nouvelles qui comprennent un nombre important

par commune déléguée. Un tel dispositif garantira une bonne représentation des communes déléguées, mais permettra aussi de s’assurer que le nombre de conseillers municipaux soit assez élevé pour répartir la charge de travail pesant sur les élus du fait de l’augmentation du périmètre communal. En particulier, cela permet de disposer d’un nombre suffisant de conseillers pour siéger dans tous les organes et commissions au sein desquels ils doivent représenter leur commune.

cela a été dit, l’application du droit commun à compter du second renouvellement général aboutit actuellement à un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. Il s’agit ici de donner la possibilité de désigner un élu supplémentaire par commune déléguée pour les communes nouvelles comprenant un nombre important de communes historiques.

historiques ou à l’origine de la création de la commune nouvelle.

monsieur les rapporteurs,

parce que la loi limite leur représentation à une personne. Or, dans la situation actuelle, force est de constater qu’une majorité des maires sont des hommes, et nous n’avons pas le pouvoir ici de décider que la moitié des communes aura une femme comme maire. Nous ne pouvons,

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.

Quel est l’avis de la commission ?

afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.